est à Mme la ministre. Si l'on veut que le raccordement électrique soit possible rapidement dès lors qu'un résident le souhaite, il est nécessaire que le pré-équipement ne se limite pas aux gaines électriques ; par exemple, les compteurs doivent être dimensionnés de manière suffisante. C'est pourquoi nous proposons de préciser que le pré-équipement comprend les dispositifs nécessaires, hors câblage, pour faciliter économiquement et techniquement l'installation ultérieure des points de recharge. amendement s'inscrit dans la lignée de l'ambition de la directive sur la performance énergétique des bâtiments en énonçant une définition du pré-équipement fonctionnelle plutôt que prescriptive. Quel est l'avis de la commission ? La rédaction proposée par le Gouvernement complète utilement la définition adoptée en commission et concilie le droit en vigueur avec les obligations nouvelles prévues par le droit européen en matière de pré-équipement.

élevé. Quel est l'avis de la commission ?

Cette transition ne pourra avoir lieu que si elle est accompagnée d'un développement important du réseau des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. C'est pourquoi je propose de doubler l'obligation : deux points de recharge

précéder la mise en place de telles obligations d'une concertation avec l'ensemble des parties prenantes- gestionnaires de réseau, promoteurs immobiliers, installateurs et représentants des copropriétés -et que le dispositif fasse l'objet d'expérimentations permettant d'en évaluer l'impact avant toute généralisation. Mme la ministre.

ne se limitent pas à l'optimisation des réseaux gaziers, mais relèvent également de l'organisation des transports. Au regard de ces enjeux multiples, un encadrement de la mesure par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie me semble préférable.

agricole. Mon département abrite le pionnier français de la méthanisation : Francis Claudepierre, qui, dès 2005, a lancé la première installation française. Aujourd'hui président de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, il m'a alerté sur le décret en cours d'écriture visant à favoriser le développement du gaz naturel végétal et de la distribution du gaz naturel. Dans le cadre de la

un développement important en France, notamment sur le marché des camions, des autobus et des autocars. Il est indispensable de continuer le soutien à cette filière, et le GNV doit être reconnu comme une réponse pertinente aussi pour les véhicules légers, en complément des véhicules électriques et hybrides. S'inscrivant dans l'esprit du projet de loi, qui vise un développement plus rapide des carburants alternatifs, la mobilité gaz terrestre pour les particuliers représente ainsi une véritable alternative dans les territoires ruraux et périurbains. Sa grande autonomie, le coût d'achat désormais proche de celui des véhicules classiques et le coût du carburant, inférieur de 20 à 30 % à celui des carburants classiques, en font un vecteur de mobilité propre très intéressant et abordable, adapté aux besoins des Français.

l'étude d'impact du projet de loi souligne que cette alternative est « un moyen d'action pour la transition énergétique permettant la maturation d'une filière plus vertueuse que le pétrole et qui a vocation à évoluer vers le bioGNV afin de répondre à nos engagements sur le climat mes chers collègues, je vous propose d'insérer le déploiement de points de recharge et de stations d'avitaillement en gaz naturel liquéfié ou comprimé à l'article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales.

permettra de réduire drastiquement notre consommation d'énergies fossiles tout en connaissant de nombreuses applications, dans les véhicules individuels comme dans les transports publics. En la matière, les technologies sont prêtes ; le seul inconvénient qui subsiste est leur prix, il est vrai encore assez élevé, mais qui baissera au fil des années, à la faveur des effets de seuil. Le présent amendement vise à inscrire dans la loi un objectif de 1 000 bornes de recharge à hydrogène à l'horizon de 2028, notamment pour contribuer à rattraper le retard important que la France a pris dans ce domaine. Certains allemands font déjà circuler des trains à hydrogène, en collaboration

représente un levier important pour la transition du secteur des transports, en particulier du transport routier et du transport fluvial. En effet, les véhicules électriques à batterie et à hydrogène limitent la dépendance à l'égard du pétrole, contribuent à la décarbonisation du secteur et atténuent l'impact environnemental des déplacements. Leur développement requiert une implication de l'État et des collectivités territoriales. De même, il est nécessaire d'assurer une visibilité aux entreprises, afin de faciliter les investissements dans la technologie des véhicules propres. L'article 41 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé l'objectif d'au moins 7 millions de points de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables d'ici à 2030. Le présent amendement tend à compléter cet objectif par un déploiement de stations de recharge à hydrogène, en cohérence avec les cibles du plan de déploiement de l'hydrogène. Cette mesure répond à la nécessité de diversifier le mix énergétique du parc automobile la complémentarité d'usages entre les véhicules électriques, adaptés aux trajets courts, et les véhicules à hydrogène pour les plus longues distances.

Personne n'est contre le développement de l'hydrogène comme solution énergétique. Mais, face à la vision idéaliste, un peu mythique, de telle ou telle solution absolument merveilleuse, qui réglera tous

l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques,- un très bon rapport n'est-ce pas, monsieur Sido ? -fait mention d'une diversité, d'un mix de solutions pour parvenir à la neutralité carbone en 2050 l'objectif fixé, en son temps, par Nicolas Hulot, alors ministre de la transition écologique, de faire cesser la commercialisation des véhicules émettant des gaz à effet de serre, les véhicules thermiques- une petite nuance qu'il avait apportée

du véhicule électrique. Si la batterie est rechargée en Allemagne, l'origine de l'énergie, c'est le lignite. Concernant le véhicule à hydrogène en France, l'hydrogène provient du craquage du méthane,

dresse toute une liste d'usages possibles dans le domaine de la mobilité. Je le redis, j'y suis évidemment favorable. D'ailleurs, depuis mon arrivée à la tête de ce ministère, nous sommes passés de 5 % des certificats d'économies d'énergie

mais aussi la consommation d'énergies fossiles. Du reste, le programme Advenir, qui soutient l'installation de bornes de recharge électrique, en est déjà une illustration, mais celle-ci est trop isolée, puisqu'il s'agit bien d'utiliser les certificats pour substituer de l'énergie décarbonée à des carburants fossiles. Si l'on veut parvenir à la neutralité carbone, il faudra mobiliser tous les outils disponibles, dont ces certificats, sachant que le secteur des transports sera le plus difficile à décarboner. il existe certes quelques programmes et fiches d'opérations standardisées dédiés à la mobilité, mais j'observe que les fiches existantes concernent uniquement des équipements et des services de niche, tels que le transport intermodal rail-route, les barges fluviales, les groupes frigorifiques, etc. Aucune ne porte, par exemple, sur des marchés de masse, tels que l'acquisition d'autobus ou d'autocars électriques ou roulant au GNV, voire à l'hydrogène. Or si l'on veut accélérer la transition énergétique dans le secteur des transports et des mobilités, il convient d'accompagner

de ce texte : pas de financement des infrastructures, aucune aide aux collectivités locales. Aussi, la commission, sous l'impulsion de son rapporteur, a proposé différents dispositifs, que M. Mandelli a rappelés précédemment, à savoir le versement mobilité à taux réduit, une part de la TICPE à destination des territoires pour lesquels le versement mobilité ne suffirait pas.

du secteur des transports ; telle n'était évidemment pas mon intention. Comme je l'ai expliqué, on est passé de 5 % seulement des certificats d'économies d'énergie utilisés au profit du secteur des transports à 12 %. Ainsi, 130 millions d'euros seront consacrés, au cours des deux prochaines années, à la mobilité. Je dis simplement que

des CEE. La loi portant engagement national pour l'environnement a étendu le dispositif aux carburants. Il se trouve que le GPL est le seul carburant alternatif concerné par ce dispositif. Les conditions du marché et la complexité de mise en oeuvre du dispositif fragilisent les entreprises de ce secteur. En effet, le marché du GPL est en décroissance de 10 % depuis cinq ans. Le réseau, bien que suffisamment développé, est fragile. Ce mécanisme accroît la pression sur la filière, qui continue d'investir, en particulier dans le développement du bioGPL. Dans le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie 2019-2023, le Gouvernement fixe l'objectif de développer le carburant alternatif GPL et le bioGPL. Par cohérence et afin de soutenir le développement de ce carburant alternatif, il semble nécessaire de l'exclure du calcul des obligations liées Cet amendement vise par conséquent à demander l'exclusion du GPL utilisé comme carburant du dispositif des CEE et, d'une manière générale, les carburants alternatifs dans leur ensemble. Le cadre fixé par la directive 2012/27/UE permet aux États membres de ne pas imposer cette obligation aux distributeurs d'énergie de petite taille, aux petites entreprises de vente d'énergie au détail et aux petits secteurs énergétiques, afin que ces derniers ne subissent pas une charge administrative disproportionnée. Quel est l'avis de la commission ? La réduction du périmètre des obligés, pour ce qui concerne les carburants, aux seuls vendeurs d'essence et de gazole remettrait en cause le principe d'universalité des certificats d'économies d'énergie, qui concernent l'ensemble des vendeurs d'énergie, quelle qu'elle soit.

est à M. Charles Revet. Les objectifs d'amélioration de la qualité de l'air et de réduction des émissions de CO2 ne pourront être atteints que par la diversification du mix énergétique et le développement de toutes les énergies alternatives. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dans son article 37, définit les véhicules à faibles émissions « comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret ». Ces critères sont restrictifs. Ils limitent la définition aux véhicules électriques et à hydrogène, laissant de côté les autres carburants alternatifs, tels que le GPL, ce qui diminue donc la portée de la mesure pour atteindre les objectifs fixés. Dans ce contexte, nous proposons de remplacer la notion de « véhicules produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques » par celle de véhicules « qui utilisent un carburant alternatif tel que défini par la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs l'avis de la commission ? L'élargissement proposé ne peut être retenu : en visant tous les carburants alternatifs au sens du droit européen, y compris, par exemple, les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques, et, surtout, en supprimant toute exigence quant au niveau des émissions de gaz à effet de serre, reviendrait à vider de sa substance la définition des véhicules à faibles émissions. Je le rappelle, cette définition concerne aujourd'hui les véhicules émettant moins de 60 grammes, et c'est ce plafond qui donne tout son sens, notamment, aux obligations de verdissement des flottes, dont nous débattrons en examinant les amendements suivants. En conséquence, je demande le retrait de cet

L'administration, les entreprises et les loueurs de véhicules représentent aujourd'hui 50 % des achats de véhicules légers neufs. La part d'achat des véhicules à faibles émissions par ces acteurs est encore très faible, contrairement à celle des véhicules diesel, encore largement majoritaire- 85 % contre moins de 20 % pour les particuliers. Ce constat va à l'encontre de l'urgence climatique et de la nécessité de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports selon une trajectoire cohérente avec les engagements climatiques de la France et comme nous le demandent beaucoup de nos concitoyens. de 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a déjà introduit des quotas de renouvellement de flottes dans une proportion minimale de 50 % de véhicules à faibles émissions pour l'État et ses établissements publics et de 20 % pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour les entreprises nationales. Nous demandons aujourd'hui que le secteur privé prenne, lui aussi, ses responsabilités environnementales. Le présent amendement vise donc à compléter le code de l'environnement, en indiquant que les entreprises du secteur privé, lorsqu'elles gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions. Cette obligation applicable immédiatement nous semble pertinente avec les enjeux liés à la qualité de l'air et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre les dérèglements climatiques.

seules les entreprises gérant un parc de plus de cent véhicules seront concernées, la plupart ayant d'ailleurs d'ores et déjà commencé à convertir leur flotte. Seuls les véhicules de moins de 3,5 tonnes seront visés, ce qui exclut le transport routier de marchandises, dont chacun connaît l'équilibre économique précaire.

pour les flottes publiques de plus de vingt véhicules automobiles, ainsi que pour les loueurs de véhicules, les taxis et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur. Les véhicules à faibles émissions sont définis comme des véhicules électriques, des véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions d'émissions de gaz à effet de serre, fixés à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette proportion de véhicules propres est fixée à 20 % pour les collectivités et leurs groupements, ainsi que pour les entreprises nationales, et à 50 % pour l'État et ses établissements publics. Pour les flottes privées, elle est fixée à hauteur de 10 % avant 2020. Afin de viser des objectifs cohérents et ambitieux de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, le présent amendement vise à rehausser la part minimale de véhicules à faibles émissions dans les parcs de véhicules d'entreprise

ainsi d'ailleurs qu'aux véhicules de gendarmerie et de police, notamment tous ces camions que l'on voit défiler dans les avenues de Paris chaque samedi

comme des voitures particulières et des camionnettes, dont les émissions de gaz à effet de serre sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone. En revanche, ce décret ne définit aucun seuil d'émission de polluants atmosphériques et ne permet pas au dispositif de viser des objectifs en termes de qualité de l'air. Ce même décret définit cependant la catégorie des véhicules à très faibles émissions comme des voitures particulières et camionnettes dont la source d'énergie repose sur l'électricité et/ou l'hydrogène. les véhicules électriques à batterie et à hydrogène n'émettent ni gaz à effet de serre ni polluants atmosphériques, et constituent des technologies complémentaires pour le déploiement à grande échelle d'un parc de véhicules propres. Nous souhaitons encourager à compter de 2021 le développement des mobilités « zéro émission » en instaurant un sous-objectif dédié aux véhicules à très faibles émissions au sein des parcs de véhicules à faibles émissions acquis ou nouvellement utilisés par les pouvoirs publics. Nous proposons que la part des véhicules à très faibles émissions soit fixée par décret. Cette mesure permettra d'anticiper la transposition de la directive relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, en cours de révision, qui prévoit de renforcer les quotas de véhicules « zéro émission » dans le cadre des marchés publics.

En effet, si les seuils fixés par les pouvoirs publics en matière de véhicules à faibles émissions traduisent une ambition qu'il faut saluer, les textes sont pour le moment assez discrets sur la question des véhicules à très faibles émissions,

l'année 2017, les ventes de véhicules électriques ont atteint 1,2 million d'unités dans le monde, soit une augmentation de près de 60 % par rapport à 2016. Le présent amendement prend en compte le coût encore relativement élevé de ces technologies et ne vise pas un objectif disproportionné. en effet à intégrer une sous-proportion de véhicules à très faibles émissions dans les parcs de véhicules à faibles émissions, avec des critères déterminés par décret. L'administration disposerait ainsi de souplesse et de temps pour anticiper les nouveaux besoins en la matière. Quel Je suis d'accord avec les auteurs de ces amendements pour considérer que les collectivités territoriales, comme l'État, doivent être exemplaires en la matière. Cela étant, le Sénat n'a pas pour vocation de créer des obligations qui pourraient être considérées comme exorbitantes.

par exemple. En renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer cette proportion minimale, le législateur renoncerait en outre à sa compétence et laisserait au Gouvernement le loisir de déterminer les obligations applicables, par exemple, aux collectivités territoriales.

Les conditions de ce remboursement sont définies à l'article 265 du code des douanes. Pour atteindre les objectifs environnementaux et sanitaires de l'État, il convient d'orienter les incitations pour encourager l'adoption de solutions alternatives et le développement d'un parc moins polluant. Cet amendement a pour objet d'inciter les taxis à utiliser le gaz de pétrole liquéfié, le GPL, en élargissant à ce carburant le remboursement d'une fraction de la TICPE. Le GPL est une solution facile à adopter pour réduire les émissions de CO2 et de polluants locaux. Dans des conditions réelles de circulation, un véhicule GPL n'émet pratiquement pas de particules. Il contribue ainsi aux objectifs fixés en matière d'amélioration de la qualité de l'air et de réduction d'émissions de CO2.

La filière aéronautique française est confrontée à un enjeu de taille : faire face au doublement du trafic prévu dans les trente prochaines années, tout en luttant contre le changement climatique. Or, parmi les différentes solutions qui ont émergé pour un transport aérien plus respectueux de l'environnement, les biocarburants sont une solution incontournable. Le Gouvernement l'a d'ailleurs reconnu en s'engageant à mettre en place une filière biokérosène en coopération avec Air France, Airbus, Safran, Suez et Total. La France a en effet un rôle primordial à jouer. Les grands groupes évoqués, tout comme les start-up françaises innovantes, proposent des solutions complémentaires pour développer ce marché, contribuer à verdir le transport aérien et à créer des emplois. amendement vise à ne pas mettre de côté le transport aérien et à poursuivre la dynamique engagée, en demandant au Gouvernement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, de remettre au Parlement un rapport sur les modalités pratiques d'un programme de soutien public pour l'émergence de filières françaises de biocarburant aéronautique. L'amendement

Or, parmi les différentes solutions qui ont émergé pour un transport aérien plus respectueux de l'environnement, les biocarburants font maintenant figure de solution incontournable. Le Gouvernement a d'ailleurs lancé une feuille de route française pour les biocarburants aéronautiques. La mise en place d'un mécanisme de soutien à la demande, pour assurer l'émergence d'un marché pérenne, est bien identifiée comme une condition nécessaire à ce développement. La France a un rôle primordial à jouer dans ce domaine. De grands groupes, comme des start-up françaises innovantes, proposent des solutions complémentaires pour développer ce marché et contribuer au verdissement du transport aérien. dans des zones rurales, permettraient de créer des centaines d'emplois, d'assurer des débouchés pour les résidus des industries agricoles et forestières ou de la biomasse ligno-cellulosique, et de revitaliser ainsi une partie de nos territoires. Nous serions aussi en phase avec les principes de l'économie circulaire en faisant en sorte d'approvisionner directement plusieurs aéroports depuis des usines de proximité. Les défis sont nombreux et les acteurs économiques ont besoin de confiance pour continuer à investir et bâtir ces usines capables de fournir les quantités suffisantes de biocarburants.

pour laquelle nous disposons aujourd'hui de très peu de leviers d'intervention, si l'on excepte des solutions à plus long terme telles que les avions solaires. Avec la mise en service d'appareils de moins en moins consommateurs d'énergie, le développement de carburants alternatifs aux carburants fossiles est certainement l'une des pistes à explorer.

quelle que soit la croissance du trafic aérien. Par ailleurs, il existe un marché ETS- -marché du carbone à l'échelle européenne, qui vise aussi à maîtriser les émissions de gaz à effet de serre dans ce secteur.

Sido, pour explication de vote. Je remercie mes collègues d'avoir maintenu leurs amendements, ce qui me permet de prendre la parole, que je demande depuis quelque temps ! J'ai essayé d'expliquer qu'il y avait électricité et électricité, hydrogène et hydrogène.

du petit nombre de rapports que l'on demanderait. Cela fait partie des sujets sur lesquels on a besoin de comprendre les grands enjeux, aujourd'hui, en termes quantitatifs. En effet, Corsia

intéressants sur la méthanisation : à partir du moment où l'on utilise les déchets agricoles, cela peut rendre quelques services. Mais se lancer en disant que, par le biocarburant,

plus fort que ce qui existe à l'échelle mondiale. Ensuite, le travail qui est en cours doit viser à ne pas demander des différents, sur la base d'indicateurs différents, aux compagnies aériennes pour répondre

concernant les gaz à effet de serre. Si ! Mis à part pour l'aviation, où des progrès pourraient être réalisés sur les motorisations et sur les masses des avions, puisqu'il faudra une certaine quantité d'énergie pour les

Depuis le début de ce quinquennat, les déceptions sur les questions environnementales ont été nombreuses. En attestent notamment la démission du ministre Hulot et le départ de Matthieu Orphelin du groupe LREM. Il faut le reconnaître, nous sommes bien loin du slogan tapageur d'Emmanuel Macron, qui déclarait voilà un peu plus d'un an plus d'un an : « » Après les reculades sur l'usage du plastique et des pesticides, après les lois Élan et Égalim, après le projet Montagne d'or en Guyane, il est vrai que nous n'attendions plus grand-chose de la part de cet exécutif. Pire encore, il y a peu, alors que se tenait la la « Marche du siècle », votre majorité parlementaire décidait de voter le report de cinq ans de l'interdiction du glyphosate. Pourtant, force est de constater que, pour une fois, le mécanisme proposé est intéressant. Loin de l'écologie inflexible et punitive, le forfait retenu semble plutôt adéquat, afin de procéder à un progressif changement, en matière de recours aux transports, vers une mobilité plus solidaire et écolo-compatible.

le principe pollueur-payeur, en rendant plus cher ce qui pollue. Vous conviendrez avec moi que ce conseil ne relève pas d'une officine de propagande révolutionnaire, puisque c'est une instance qui travaille pour le Premier ministre. CAE envisage donc un chèque énergie et un principe de redistribution très fort pour relancer cette mécanique vertueuse, ce qui va tout à fait dans le sens de la proposition de loi sur le pouvoir d'achat

L'article L. 3261-2 du code du travail prévoit quant à lui que l'employeur prenne en charge une partie du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen d'un service public de location de vélos. Cet amendement tend à étendre cette prise en charge par l'employeur aux services privés de location de vélos lorsqu'il n'existe pas d'offre publique, et ce pour développer les mobilités actives. Quel monsieur le rapporteur,

mettre en place un forfait mobilités durables exonéré de charges sociales et de charges fiscales. J'ai eu l'occasion de le dire, des discussions sont en cours avec les partenaires sociaux, et en particulier avec les employeurs, pour voir comment nous pouvons aller plus loin-

de travail est une bonne façon d'encourager l'utilisation des véhicules électriques. Aujourd'hui, dans le cadre réglementaire actuel, un employeur qui met à disposition de ses salariés une recharge gratuite

à la prise en charge obligatoire du forfait mobilités durables par les entreprises, pour les salariés qui connaissent des difficultés dans leur trajet domicile-travail. Vous avez raison : les Français

afin de prendre en charge tout ou partie de leurs frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail, à vélo ou en tant que passager en covoiturage. Nous souhaitons, comme M. Bonhomme, rendre ce

Cette modification est cohérente avec l'obligation déjà faite à l'employeur de prendre en charge une partie des abonnements de transports publics souscrits par ses salariés,

? On peut décider de consacrer son temps à se transporter : c'est très bien, mais c'est très cher, car le temps perdu ne se retrouve jamais !

mesure une seule enveloppe globale portée à 600 euros par an. Il tend également à permettre le défraiement par les entreprises des modes de transport utilisés par les salariés dans leurs déplacements domicile-travail frais de transport public, de transport personnel, de carburant ou d'alimentation électrique et de dépollution du véhicule, avec la possibilité de combiner ces usages à tout moment. Les

de rembourser à leurs salariés une partie de leurs frais de déplacement domicile-travail, sous réserve de l'utilisation d'un mode vertueux de transport, comme le vélo ou le covoiturage. Cette enveloppe représente assurément un formidable levier de facilitation et de développement des mobilités responsables.

tout ou partie des frais engagés par les salariés pour effectuer leurs trajets domicile-travail à vélo ou en covoiturage. En ce qui concerne le vélo, le texte de l'article précise qu'il s'agit de trajets effectués à « vélo » ou à « vélo à assistance électrique Nous considérons que ce champ d'application est trop restreint et que d'autres types d'engins de déplacement personnel ou des véhicules de type nouveau, comme le vélomobile, doivent être pris en compte. Le vélomobile est un hybride entre le vélo et la voiture, que l'on conduit couché et protégé par une carrosserie aérodynamique. Il offre un nouveau mode de déplacement adapté aux trajets domicile-travail, dans la mesure où il abrite ses occupants des intempéries et peut atteindre des vitesses de l'ordre de 50 kilomètres par heure. avons de bonnes raisons de penser que l'innovation en matière de mobilité ne s'arrêtera pas au lendemain de la promulgation de cette loi. Il convient donc de ne pas restreindre le forfait mobilités durables

Cet amendement est dans la même veine que celui qui vient d'être évoqué, il vise à ne pas limiter le forfait mobilités durables au vélo personnel et au covoiturage, et donc à y intégrer d'autres modes de transport propres ou partagés, comme le vélo en libre-service et les trottinettes personnelles ou en libre-service.

tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo ou vélo à assistance électrique personnel [ ...]. » Je vous fais grâce du covoiturage,

n° 369 rectifié. L'article 26 du projet de loi crée un forfait mobilités durables facultatif permettant aux entreprises et aux administrations de rembourser à leurs salariés et agents une partie de leurs frais de déplacement domicile-travail. Ce forfait s'applique aux modes de déplacement permettant de réduire la pollution, comme le vélo ou le le covoiturage. C'est une politique incitative qu'il convient de saluer, par opposition à une écologie punitive. Le forfait, d'un montant maximal de 400 euros, est exonéré de charges sociales et d'impôt sur le revenu. Chaque salarié pourra choisir chaque mois de bénéficier du forfait mobilités durables, d'être couvert par la prise en charge d'une partie de l'abonnement pour les transports collectifs, ou de continuer à percevoir le remboursement des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, dans la limite de 200 euros par an. amendement vise à ajouter la recharge d'hydrogène au mode d'alimentation pris en compte par ce dispositif et à introduire une distinction entre carburants vertueux sur le plan environnemental et carburants fossiles, en étendant le bénéfice des 400 euros du forfait mobilités durables aux frais d'alimentation des véhicules électriques et à hydrogène.

permettant de réduire la pollution comme le vélo ou le covoiturage. Le forfait, d'un montant maximal de 400 euros, est exonéré de charges sociales et d'impôt sur le revenu. Chaque salarié pourra choisir chaque mois de bénéficier du forfait mobilités durable, d'être couvert par la prise en charge d'une partie de l'abonnement pour les transports collectifs, ou de continuer à percevoir le remboursement des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, dans la limite de 200 euros Le présent amendement vise à introduire une distinction entre carburants vertueux sur le plan environnemental et carburants fossiles, en étendant le bénéfice des 400 euros du forfait mobilités durables aux frais d'alimentation des véhicules électriques à batterie et à hydrogène. Ce montant resterait de 200 euros pour ce qui relève du remboursement des frais de carburants. Dès lors, ce dispositif d'aide par l'employeur doit permettre d'encourager le développement de la mobilité propre, en cohérence avec l'objectif de lutte contre la pollution de l'air visé par le présent article, avec, d'un côté, un forfait mobilités durables couvrant la mobilité active et partagée et, de l'autre, la mobilité zéro émission concernant l'électricité et l'hydrogène. La parole

L'objet du présent amendement est d'étendre le bénéfice des 400 euros du forfait mobilités durables aux frais d'alimentation des véhicules électriques et à hydrogène. Ce montant resterait de 200 euros pour ce qui relève du remboursement des frais de carburants.

est à Mme la ministre. Votre commission a proposé de rendre possible le cumul du forfait mobilités durables avec la prise en charge par l'employeur d'une partie des frais d'abonnement de ses salariés aux transports publics ainsi que de leurs frais de carburant, et ceci, sans poser de conditions particulières. Il me semble très important que les employeurs accompagnent la mobilité de leurs salariés et encouragent le développement des mobilités actives et partagées,

et vise à revenir à la rédaction initiale du projet de loi, lequel prévoyait le versement d'une prime de façon volontaire par les entreprises. Il faut rappeler que les entreprises financent largement le transport des salariés avec le versement transport et la participation au remboursement des frais de déplacement en transports collectifs. Rendre obligatoire le cumul de ces dispositifs avec le forfait mobilités durables emportera de lourdes conséquences financières, notamment pour les petites et moyennes entreprises. maintenir le caractère volontaire et non cumulable du forfait mobilités durables. L'amendement

936 et 430 rectifié ? En commission, nous avons adopté un amendement visant à permettre aux salariés de bénéficier, au titre d'un même mois, du cumul entre le forfait mobilités durables et la prise en charge par l'employeur d'une partie de leurs frais de transport en commun.

actives. Quel est l'avis de la commission ?

des abonnements de transports en commun. En effet, il faut éviter de détourner des transports de personnes les salariés qui pourraient, par une prise en charge nouvelle, faire d'autres choix de mobilité. Le pouvoir réglementaire avait fixé à 50 % le niveau de prise en charge du prix des titres d'abonnement par l'employeur. Une étude de l'Insee sur les déplacements des salariés en 2015 montre que 63 % des cadres et 65 % des employés utilisent la voiture pour leurs déplacements professionnels, contre 75 % pour les professions intermédiaires et 78 % pour les ouvriers, notamment en raison des coûts de transport. Dès lors, afin de favoriser significativement les déplacements en transports en commun, nous proposons, avec cet amendement, que les employeurs prennent en charge intégralement, et non plus à moitié, les frais d'abonnement de leurs salariés. Une telle mesure serait un signe fort pour réorienter les salariés de la voiture individuelle vers les transports collectifs, lorsque ceux-ci existent, bien sûr. Ainsi, les salariés pourront favoriser les transports collectifs tout en gagnant en pouvoir d'achat, tandis que les employeurs seront davantage associés aux efforts pour la mobilité propre en étant sensibilisés au développement des transports collectifs.

des salariés au SMIC. Dans le budget des ménages, les transports représentent le premier pôle de dépenses devant le logement. Dès lors, la prise en charge intégrale des frais de transport professionnels pour les personnes au SMIC serait une mesure de justice sociale. Gontard. Il nous paraît indispensable de rendre cumulables la prise en charge partielle par l'employeur d'un abonnement de transports collectifs et celle d'un abonnement de service de location de vélos pour favoriser l'intermodalité. Les usagers du vélo sont nombreux à utiliser les transports en commun, et vice-versa, qu'il s'agisse d'un même trajet ou simplement de différentes périodes de l'année, pour éviter, par exemple, le vélo les jours de pluie. Il convient d'encourager cette complémentarité entre des modes de transport vertueux. Par ailleurs, Par ailleurs, il arrive à de nombreuses personnes de combiner vélo et transports en commun pour un même trajet. Cette mesure est donc également une incitation à la multimodalité, qui est prônée par ce projet de loi. de la prise en charge d'un abonnement à un service de location de vélos à l'année, de l'ordre de quelques dizaines d'euros, est marginal pour les entreprises. Il s'agit davantage d'envoyer un message aux salariés pour les inciter à faire évoluer leur usage de mobilité vers les mobilités actives. Quel est l'avis de la commission ? Les entreprises Les entreprises prennent d'ores et déjà en charge 50 % des frais d'abonnement aux transports publics de leurs salariés. Prévoir une prise en charge intégrale représenterait

Seront notamment testées des zones à faibles émissions au sein de ces grandes métropoles. Comme pour l'article 26, l'intention est louable, mais la mesure n'est pas à la hauteur de la situation. La pollution est globale et touche et touche nos 68 millions de concitoyens. Pourtant, vous semblez privilégier l'amélioration de la qualité de l'air uniquement pour les citadins des grandes villes. Allons-nous, une fois de plus, feindre d'oublier que plus de 20 % de la population vit encore en zone rurale ? Allons-nous ignorer également les derniers rapports démographiques de l'Insee, selon lesquels ce sont les villes de 10 000 à 50 000 habitants qui connaissent la plus forte expansion ? À la fracture sociale et économique qui sépare aujourd'hui nos grands centres urbains de nos campagnes va-t-on ajouter une fracture sanitaire ? En partant de ce constat, il est évident que ce seuil de 100 000 habitants n'est ni suffisant ni ambitieux. Ce manque d'inspiration est également illustré par le temps long que s'accorde l'exécutif pour mettre en place les dispositifs. Si vous me permettez de reprendre la fameuse expression de Jacques Chirac, « la maison brûle », et nous attendons l'horizon 2025-2030 pour agir. La transformation du secteur des transports est urgente et incontournable pour respecter les engagements pris dans le cadre de la COP 21. Vous avez l'occasion d'enclencher cette transition, tout en apportant des solutions aux difficultés auxquelles nos concitoyennes et concitoyens sont confrontés au quotidien. Ayez l'audace de proposer de véritables mesures novatrices, comme la gratuité des transports en commun qui aurait pour mérite de désengorger les réseaux routiers, tout en améliorant durablement la qualité de l'air. C'est vers cela que doit tendre la mobilité du XXI siècle.

sont les outils privilégiés des collectivités territoriales pour anticiper et préparer la transition écologique. Par ailleurs, cet article prévoit que les plans d'action de lutte contre la pollution de l'air devront permettre d'atteindre, à compter de 2025 et 2030, des objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national. Nous proposons de supprimer cet échéancier qui n'apporte aucune valeur ajoutée aux dispositions prévues

d'un plan d'action pour la réduction des taux de concentration de polluants atmosphériques en ciblant particulièrement les zones à proximité des établissements recevant un public sensible, comme les établissements d'accueil des jeunes enfants, les écoles, les structures d'hébergement des personnes âgées, les hôpitaux, les équipements sportifs et les espaces extérieurs dédiés aux activités sportives, et ce d'ici à 2025.

Obliger tous les EPCI de plus de 50 000 habitants à inclure dans leur PCAET des plans de lutte contre la pollution de l'air me paraît trop contraignant et risque de retarder encore davantage l'adoption de ces plans. L'avis est défavorable. En ce qui prévoir que les taux de concentration auxquels sont exposés les établissements recevant un public sensible doivent être inférieurs aux valeurs limites de pollution de l'air recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, est souhaitable. Mais, avant de respecter ces niveaux, encore faudrait-il commencer par respecter les normes prévues par le droit européen. Je vous rappelle que la France fait l'objet d'un contentieux au niveau européen, puisque la Commission européenne a saisi le 11 octobre dernier la Cour de justice de l'Union européenne pour non-respect des valeurs limites de dioxyde d'azote. L'avis est également défavorable. Quel est

Diminuer les problèmes de pollution, cela ne se fait pas d'un claquement de doigts, sinon on se demande bien pourquoi cela n'a pas été fait jusqu'à présent. Je pense qu'il n'est pas du tout réaliste d'imposer que ces objectifs soient atteints d'ici à 2020, même si, bien évidemment, il est souhaitable qu'ils le soient au plus tôt. Je propose donc le retrait des

Lamure. L'article 27 du projet de loi prévoit que les EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants ou dont le territoire est couvert par un plan de protection de l'atmosphère établissent des plans d'action de lutte contre la pollution de l'air. Il est prévu que ce plan d'action comporte obligatoirement une étude sur la mise en place d'une ou plusieurs zones à faibles émissions, ou ZFE. Cet amendement tend à supprimer cette obligation, dans le respect du principe de libre administration des collectivités locales. Il est préférable de laisser la faculté aux EPCI d'entreprendre ce type d'études très coûteuses sans les y contraindre, sauf à prévoir une compensation financière pérenne, ce qui ne semble pas être le cas dans le projet de loi.

L'article 27, qui fait l'objet de cet amendement, impose d'élaborer une étude portant sur la mise en place d'une zone à faibles émissions dans le cadre des plans d'action de lutte contre la pollution de l'air. Nous ne sommes pas opposés à la mise en place de telles zones, qui contribuent à l'objectif de lutte contre la pollution de l'air. Cependant, nous souhaitons que, dans le cadre de ces zones, les éventuelles restrictions de circulation des voitures soient corrélées à la mise en oeuvre de la gratuité des transports lors des pics de pollution. Si des mesures ont déjà été mises en place afin d'inciter les automobilistes à ne pas utiliser leur véhicule, comme la gratuité des covoiturages ou du stationnement résidentiel pour les Parisiens, elles sont, à notre avis, insuffisantes. C'est également la position de la mairie de Paris, qui a appelé, il y a quelques mois, le Gouvernement à agir, notamment en demandant la gratuité des transports publics en Île-de-France. L'interdiction de la circulation des véhicules automobiles lors des pics de pollution est une solution efficace et inévitable. Cependant, si l'on veut que nos concitoyens puissent la respecter, il est nécessaire de leur en donner les moyens et de proposer un mode de transport alternatif. Les automobilistes ont des frais fixes liés à l'utilisation de leur véhicule, comme le coût d'achat, l'entretien ou encore les frais d'assurance. Leur imposer d'utiliser les transports en commun ne doit pas engendrer de frais supplémentaires. Enfin, vous le savez, la gratuité des transports en commun est une revendication de longue date de notre groupe : cette gratuité doit être permanente, et pas seulement lors des pics de pollution. telle mesure a des effets positifs, comme l'ont montré les expérimentations déjà menées dans une vingtaine de communes françaises. Je suis sûr que la mission d'information sur cette question, dont fait partie notre collègue Guillaume Gontard, le démontrera. Nous aurons l'occasion d'en discuter

de 2025 à 2020 la date à partir de laquelle ils pourront étudier les solutions sur les véhicules à zéro émission moteur. Il s'agit d'un amendement incitatif

permettant de lister toutes les initiatives en matière de mobilité verte en France. On peut donc imaginer que cette mesure permettra le partage d'idées et de bonnes pratiques, ce qui justifie de prendre de l'avance sur les véhicules à zéro émission moteur.

de mettre en oeuvre la gratuité dans les transports lors des pics de pollution a en effet assez peu de rapport avec les ZFE, qui visent une action de fond. Je rappelle que, lors de tels pics, il

qui contient déjà un plan d'action intitulé en ces mêmes termes. Les objectifs globaux du PCAEM, et donc de son plan d'action, sont le respect des normes en matière de polluants en 2024 et des objectifs de l'OMS en 2030. Le plan d'action prévoit l'accompagnement à la création d'une ZFE métropolitaine, pour l'action AIR3. Cependant, l'étude de préfiguration de la ZFE n'est pas intégrée au plan d'action du PCAEM, mais tirée à part. Ainsi, le PCAEM répond sur le fond aux exigences posées par l'article 27 du projet de loi. Le présent amendement a pour objet d'éviter à la métropole du Grand Paris, ou à toute autre collectivité susceptible de se trouver dans la même situation, de réviser son PCAEM pour une question de forme uniquement, à savoir

En effet, la législation en vigueur « engendre » des PPA qui peuvent concerner une seule commune d'une intercommunalité, comme c'est actuellement le cas dans l'agglomération de Nancy. De telles situations sont paradoxales, alors que les intercommunalités ont un rôle à jouer dans la mise en oeuvre du PPA, notamment lorsqu'elles possèdent la compétence de lutte contre la pollution de l'air. En permettant que toute l'intercommunalité soit, dans un délai maximal de cinq ans, rattachée au plan de protection de l'atmosphère qui concerne à l'origine seulement une partie de son territoire, le présent amendement permet, dans un souci de cohérence et d'efficacité, d'améliorer l'implication de l'intercommunalité dans la mise en oeuvre du PPA.

les EPCI ayant déjà réalisé une étude de préfiguration relative à l'instauration d'une ZFE ne se voient obligés d'en faire une nouvelle, compte tenu des dispositions du projet de loi. Toutefois, il me semble- Mme la ministre pourra peut-être le confirmer -que la rédaction de l'article 27 permet déjà d'exclure de cette obligation les EPCI ayant déjà réalisé une étude sur la mise en place d'une ZFE dans le cadre de leur PCAET.

tel qu'il est rédigé, on peut comprendre que le seul fait d'avoir engagé une étude permettrait de dispenser d'intégrer un plan d'action dans le cadre du PCAET, ce qui ne paraît pas souhaitable.

Toutefois, ce sont les préfets qui sont compétents pour modifier les plans de protection de l'atmosphère. Je ne suis pas sûr qu'une disposition législative soit nécessaire pour parvenir à cette fin.

Par ailleurs, une étude de préfiguration d'une zone à faibles émissions a été réalisée par la métropole ; cette zone est en cours de création. Les établissements publics territoriaux de la métropole élaborent, pour leur part, un

les EPT à réaliser des études relatives à des ZFE réduites à leurs territoires. Le présent amendement a donc pour objet de limiter le contenu du plan d'action des PCAET au premier alinéa du 3° 3° du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Quel est l'avis de la commission ?

Une zone à faibles émissions métropolitaine est en cours de création, sous l'impulsion de la métropole du Grand Paris. de sa création, chaque maire des communes membres de la métropole et incluses dans le périmètre de la ZFE doit édicter un arrêté concordant pour son territoire communal.

Je comprends l'objet de cet amendement, mais ce dispositif pose deux types de problèmes. Le premier problème est juridique : cette mesure reviendrait à transférer à la métropole du Grand Paris une partie des pouvoirs de police de la circulation des maires, mais non leur totalité. Cela poserait des difficultés, puisque la métropole serait compétente pour mettre en place des restrictions de circulation

aux AOM de mettre en place, à l'entrée des grandes villes, un péage positif. À contre-pied de toute logique punitive, ce dispositif permettrait de proposer à certains automobilistes d'adhérer à un programme volontaire incitatif, fondé sur une rétribution temporaire de l'évitement des heures de pointe ou du report vers des modes de déplacement plus doux. Sa finalité serait d'ancrer chez les automobilistes des habitudes durables pour limiter la congestion des axes routiers. De tels péages ont été mis en place aux Pays-Bas, en particulier, où ils ont rencontré un vif succès. La métropole européenne de Lille- vous le savez -a pour projet d'en mettre un en place. Si l'on peut comprendre la décision du Gouvernement de supprimer dans le texte toutes les mesures relatives aux péages urbains, compte tenu du contexte actuel et de la nécessité de garantir que l'écologie soit le corollaire de la justice fiscale, il est dommage qu'il n'ait pas fait preuve d'innovation et prévu les mesures nécessaires à la mise en place de péages

traversent le département sans s'arrêter. Ce trafic pourrait être aisément reporté sur l'autoroute A 10, qui est proche, puisqu'elle effectue un trajet parallèle à la route nationale entre Poitiers et Bordeaux. Les camions préfèrent circuler sur la route nationale parce qu'elle n'est pas assujettie à péage ; ils acceptent d'allonger de quelques minutes leur temps de trajet, pour une économie de bouts de chandelles Aussi, dans un souci de lutte contre la pollution atmosphérique résultant du trafic de ces poids lourds, cet amendement vise à octroyer aux maires ou aux présidents d'EPCI dont la collectivité est située à moins de 50 kilomètres d'une autoroute à péage le pouvoir d'établir une zone à circulation restreinte sur le territoire de leur commune ou de leur EPCI. Ainsi, les camions quitteront la route nationale pour l'autoroute, qui est adaptée à ce trafic et lui dédie

est ainsi libellé : La parole est à M. Éric Gold. Cet amendement vise à élargir le champ des territoires pouvant être inclus dans une zone à faibles émissions. Toutes les communes compétentes d'un EPCI pourront mettre en place une ZFE, et non pas seulement les agglomérations de plus de 100 000 habitants. permettrait d'augmenter l'attractivité des villes moyennes et de revaloriser le foncier dans leurs centres-villes grâce à une action résolue sur les mobilités durables. Par ailleurs, une étude de 2016 de Santé publique France démontre clairement que tous les territoires sont touchés par la pollution de l'air. Les centres urbains des communes moyennes n'en étant pas exempts, il convient d'agir, pour des raisons prioritaires de santé publique,

a pour objet d'élargir le dispositif des zones à faibles émissions à toutes les agglomérations comptant plus de 50 000 habitants, soit environ 80 communes et 5 millions d'habitants supplémentaires.

le seuil de 50 000 habitants pour les agglomérations existe déjà dans les outre-mer, notamment en matière de perception de la taxe spéciale sur les carburants. Toute agglomération comptant au moins 50 000 habitants peut percevoir

M. Roland Courteau. Cet amendement a pour objet d'adapter les restrictions propres aux zones à faibles émissions à certains types de publics, y compris aux plus fragiles. souhaitons ne pas sanctionner davantage des individus ne disposant pas des ressources nécessaires pour l'acquisition d'un véhicule propre ; par ailleurs, si les moyens de transport de substitution sont insuffisants ou inadaptés,

a également pour objet- c'est important -de faire en sorte que la mise en place des ZFE soit complétée par un plan d'action comportant des mesures d'accompagnement. En effet, une étude de l'Ademe de mars 2018 sur les zones à faibles émissions

monsieur le rapporteur, Je tiens à rappeler que les collectivités qui créent des ZFE disposent de larges marges de manoeuvre pour définir les voies de circulation et les catégories de véhicules concernées, ainsi que les horaires et les jours pendant lesquels les restrictions de circulation s'appliquent. Une vraie liberté est donc laissée aux collectivités pour adapter ces ZFE ces ZFE aux spécificités de leur territoire, ce qui leur permet notamment de tenir compte de l'offre de mobilité disponible. À ce titre, d'ailleurs, les collectivités peuvent accorder des dérogations individuelles pour permettre à certaines personnes de circuler dans ces zones.

d'une analyse des populations concernées par le risque de dépassement des normes de qualité de l'air, mais aussi de la proportion de véhicules concernés. Le projet d'arrêté, assorti de l'étude, est soumis pour avis à l'autorité compétente, aux autorités organisatrices de la mobilité, aux conseils municipaux

En 2030, dans onze ans, seuls les véhicules dits « propres » pourront circuler dans la zone à faibles émissions de la métropole du Grand Paris. Je m'en réjouis, d'abord, parce que l'enjeu climatique et environnemental constitue le défi à relever pour notre génération. Je m'en réjouis, aussi, parce que la mise en place de cette ZFE implique obligatoirement que le Gouvernement offre des alternatives sérieuses aux habitants de grande banlieue, qui sont aujourd'hui contraints de prendre leur voiture pour aller travailler. Je m'en réjouis, enfin, parce que je me préoccupe depuis vingt ans de la situation déplorable du réseau RER en Île-de-France. La mise en place de la ZFE obligera le Gouvernement à débloquer de gros moyens en très peu de temps pour les RER. Pour que la ZFE fonctionne vraiment et pour lutter vraiment contre la pollution, il faut augmenter vraiment la fiabilité et la régularité des RER,

Madame la ministre, peut-on imaginer mettre en place la ZFE sans offrir d'alternatives aux Franciliens ? Va-t-on abandonner davantage les habitants de grande couronne, en les privant purement et simplement d'accès à Paris ? C'est pourquoi cet amendement a recueilli les signatures de cinq groupes politiques et représentant les quatre départements de la grande couronne. Alors, de deux choses l'une, madame la ministre : soit on veut que les RER fonctionnent en 2030 de manière à permettre à la ZFE d'exister et aux habitants de la grande couronne de se rendre à leur travail dans de bonnes conditions, auquel cas nous comptons sur vous pour soutenir cet amendement, soit on sait d'ores et déjà qu'il ne sera pas possible d'offrir des alternatives sérieuses aux habitants les plus éloignés de Paris, éloignés de Paris, et on se moquera totalement de ces habitants, de leur santé, du climat et de la pollution ! Dans ce cas-là, en effet, il vous faut émettre un avis défavorable sur cet amendement, en utilisant un prétexte technique pour balayer en un instant les préoccupations de 5,5 millions de de Franciliens qui vivent en grande couronne. Mes chers collègues, les habitants de grande banlieue subissent les mêmes difficultés de déplacement que les habitants des zones périurbaines de province. Le quotidien d'un habitant de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, est plus proche de celui d'un habitant de la périphérie d'Angers, de Nîmes, ou de Tourcoing, que de celui d'un Parisien. L'objet de cet amendement dépasse largement le cadre strict de l'Île-de-France. Nous demandons simplement que les habitants des zones périurbaines soient respectés. J'en appelle donc à la solidarité et à la responsabilité de tous nos collègues issus de territoires de plus en plus ignorés

à la réalisation de lignes à grande vitesse, pour s'occuper des transports du quotidien. Je ne peux donc pas laisser dire que l'on ignore les habitants de ces zones. Tout ce que vous êtes en train de voter dans le cadre de ce projet de loi vise précisément à prendre en compte les transports du quotidien, ceux des habitants des centres-villes, des zones périurbaines, des villes moyennes, des petites villes et des zones rurales, que l'on a pendant trop longtemps ignorés. S'agissant en particulier de l'Île-de-France, j'ai émis un avis défavorable

sur les transports en commun, y compris ferrés, en Île-de-France, comme je souhaite qu'on le fasse dans toutes les grandes métropoles, qui ont pris un retard considérable

l'État et la région consacrent énormément de moyens non seulement au Grand Paris Express, qui est payé par les Franciliens et les entreprises franciliennes, mais aussi à l'amélioration du réseau existant

À Sainte-Geneviève-des-Bois, on met trois heures par jour pour aller travailler : une heure et demie à l'aller ; une heure et demie au retour. J'en parlais avec des collègues, il est plus rapide de venir du Mans

En effet, depuis plusieurs décennies, nous sommes bien obligés de constater qu'un certain nombre d'efforts qui auraient dû être faits ne l'ont pas été. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la situation que vient de décrire notre collègue Olivier

une tante qui habite Saint-Michel-sur-Orge, commune voisine de Sainte-Geneviève-des-Bois et qui a travaillé- elle est aujourd'hui à la retraite -durant toute sa carrière à Paris, à l'hôpital, où elle était infirmière. Ce que vous disiez est fort juste, elle avait droit à trois heures de transport par jour

Ce dispositif, s'il est appliqué sur de nombreux territoires, doit répondre à deux principes. Tout d'abord, une durée minimale d'application de trois ans offrira une visibilité et une prévisibilité suffisantes pour les acteurs économiques.

C'est pourquoi cet alinéa modifie le II de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

L'article 28 tend à transformer les zones à circulation restreinte en zones à faibles émissions d'ici à la fin de l'année 2020. Les interdictions de circulation des véhicules sont fondées sur leurs émissions polluantes. Leur application doit prendre en compte le calendrier des évolutions technologiques en matière de motorisation et la disponibilité du parc. Afin de permettre à chacun de programmer les investissements nécessaires au renouvellement des véhicules, il est important d'offrir de la prévisibilité prévisibilité aux acteurs de la mobilité. En effet, les interdictions ne doivent pas avoir pour effet d'interdire l'accès des TPE et PME à certains marchés.

Dans les deux cas, cela revient à encadrer la compétence des collectivités, alors que certaines pourront souhaiter créer une ZFE sur une période courte, afin de procéder à son évaluation et, si besoin, à son ajustement, lorsque d'autres collectivités envisageront

Il y a effectivement besoin de donner de la visibilité sur les mesures qui seront prises en matière de circulation. C'est le principe même des zones à faibles émissions que de mettre en oeuvre des dispositions progressives

: La parole est à M. Patrick Chaize. En l'état actuel de la législation, les émissions polluantes dégagées par les dispositifs embarqués à bord des véhicules, tels que les groupes frigorifiques disposant d'un moteur autonome, ne sont pas prises en compte pour fixer les mesures de restriction de circulation applicables au sein des zones à circulation restreinte, renommées zones à faibles émissions à la faveur du présent projet de loi d'orientation des mobilités, et déterminer les catégories de véhicules concernés au sein de ces mêmes zones. Pourtant, la majorité des groupes frigorifiques actuels produisent du froid grâce à un moteur thermique autonome. Ces moteurs produisent non seulement beaucoup de bruit, mais représentent aussi plus de 90 % des émissions de particules d'un camion frigorifique pris dans son ensemble, motorisation comprise. Pourtant, des solutions alternatives propres existent et sont d'ores et déjà déployées ; elles fonctionnent notamment à l'électricité ou à l'azote cryogénique. Afin de mieux protéger les populations exposées aux émissions de ces dispositifs embarqués et d'encourager le remplacement des solutions traditionnelles par des solutions propres, cet amendement prévoit que soit tenu compte des émissions des dispositifs embarqués lors de la détermination et de la mise en oeuvre des mesures de restriction de circulation au sein des zones à faibles émissions.

Par cet amendement, il s'agit d'associer les organisations professionnelles du secteur des transports à la concertation liée à la création des zones à faibles émissions et aux limitations de circulation dans ces zones. Les interdictions de circulation des véhicules fondées sur leurs émissions polluantes doivent être adoptées selon un calendrier tenant compte des évolutions technologiques et de la disponibilité de véhicules aux motorisations alternatives, en particulier pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes affectés au transport des personnes.

l'avis du Gouvernement ? Je pense en effet que l'association des chambres consulaires doit permettre de recueillir l'avis des entreprises, notamment les entreprises de transport routier. Par ailleurs, les collectivités pourront tout à fait associer spécifiquement des entreprises particulièrement

l'alinéa 23 de l'article 28 dispose : « Les lieux d'implantation des dispositifs fixes sont déterminés en tenant compte des niveaux de pollution atmosphérique observés sur les voies de circulation concernées. »

de la discussion des amendements précédents. Or, pour pouvoir déployer efficacement ces ZFE, les AOM doivent avoir accès à des outils de contrôle automatisé efficaces et crédibles, ce que seule l'instauration d'un vidéocontrôle peut assurer. Toutefois, l'arrêté autorisant l'installation de ces dispositifs ne peut être délivré qu'à certaines conditions strictes qui en limitent l'efficacité. Le présent amendement vise vise donc à assouplir ces contraintes. Ces assouplissements ne mettent pas à mal l'équilibre entre, d'une part, les principes constitutionnels de respect de la vie privée et de liberté de circulation

Toutefois, le déploiement des dispositifs de contrôle doit aussi veiller à ne pas porter des atteintes disproportionnées aux libertés individuelles, ce qui nécessite de trouver un compromis entre la portée des contrôles et leur proportionnalité.

que les limitations et précautions dont est assortie la procédure de contrôle étaient « de nature à assurer la conciliation qu'il incombe au législateur d'effectuer entre, d'une part, le respect de la vie privée des personnes et la liberté d'aller et venir et, d'autre part, la répression des infractions aux règles édictées dans la zone à faibles émissions

ces limitations. Toutefois, compte tenu du caractère potentiellement intrusif des dispositifs de contrôle, il est nécessaire que la loi fixe certaines limites. C'est pourquoi j'invite les auteurs de ces amendements à les retirer au profit de la solution de compromis adoptée en commission.

efficace et dissuasif au contrôle tout en respectant les droits et libertés des automobilistes. Mais, à la différence des voies réservées, qui peuvent généralement être évitées par les automobilistes, les zones à faibles émissions concernent des quartiers

L'avis du Conseil d'État est assez clair sur ce sujet : il est bien précisé que les dispositifs de contrôle automatisé de ces zones doivent être assortis de garanties spécifiques pour ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir ou à la vie privée des automobilistes. Sur la base de la définition de ces atteintes, qui ne doivent pas être disproportionnées, la commission des lois considère qu'il est indispensable d'inclure dans le texte des garanties spécifiques supplémentaires pour encadrer la mise en place du contrôle-sanction automatisé des ZFE : limitation du nombre de contrôles journaliers, absence de contrôle de l'ensemble des véhicules.

Par ailleurs, il faut évidemment que les élus qui créeront ces ZFE envisagent un processus très progressif,

fichiers. Soyons clairs : nous partageons l'idée de la mise en place obligatoire de ZFE avant le 31 décembre 2020 dans les territoires où les normes de qualité de l'air ne sont pas respectées. en revanche, moins convaincus par la possibilité créée par le présent article, pour les services de police et de gendarmerie nationales et pour les services de police municipale, de mettre en oeuvre des dispositifs de contrôle automatisé de ces zones et, une nouvelle fois, de constituer des fichiers, même périssables. Selon les termes de cet article, en effet, ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules identifiés au titre de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique, ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés.

des efforts ont été faits sur la question du contrôle d'identité : il est prévu désormais que ces contrôles devront faire l'objet d'un traitement afin de masquer de manière irréversible l'identité des passagers du véhicule et des tiers, ce qui nous semble positif. le Conseil d'État avait émis un certain nombre de réserves sur ce procédé. Il avait ainsi jugé la création d'un tel dispositif de recueil massif de données potentiellement identifiantes comme susceptible d'attenter aux principes constitutionnels de respect de la vie privée et de liberté d'aller et venir. Il avait finalement estimé, en raison du motif d'intérêt général recherché et de la nécessité de faire respecter les restrictions de circulation qui en découle, que ces mesures étaient équilibrées au regard des limitations et précautions dont est assortie la procédure de contrôle, ces limitations étant de nature à assurer la conciliation qu'il incombe au législateur de garantir entre les différents principes et intérêts en cause. L'évolution du texte en commission, le taux de

est à Mme la ministre. J'ai déjà eu l'occasion de présenter un amendement du même type à propos d'autres dispositifs de contrôle. La commission a introduit l'obligation d'un masquage irréversible des tiers et des passagers du véhicule. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, en l'état des technologies, il n'est pas possible de

pas l'atteindre aux dépens de la liberté individuelle et de la capacité de chacun de se protéger contre les excès possibles des fichiers. On crée un fichier pour quelque chose, puis on en change la finalité,

même avec l'objectif le plus digne ! On ne peut pas atteindre un objectif aussi digne que la mobilité écologique au détriment de la liberté des Français

Le Gouvernement partage l'objectif de donner des moyens aux collectivités qui mettent en oeuvre les dispositifs de contrôle. Mais, dans la pratique, plusieurs schémas seront sans doute choisis, selon les cas et les compétences des différentes collectivités. L'adaptation du dispositif général d'affectation des recettes de contrôle automatique au compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » pour le cas spécifique des zones à faibles émissions doit donc faire l'objet de réflexions et de concertations approfondies. En attendant, je vous propose de supprimer l'alinéa

le trafic automobile sur les principaux axes des grandes agglomérations françaises cause des nuisances très significatives en termes de pollution et de bruit. Si une partie de ce trafic peut être notamment réduite par le développement des transports en commun locaux, une autre part est constituée par des usagers en transit qui ne font que traverser les agglomérations, créant des problèmes de congestion et des nuisances dans des zones souvent densément peuplées. nécessaire pour ces personnes de traverser l'agglomération pour se rendre à leur destination, en particulier lorsqu'il existe des voies de contournement à forte capacité. Il faut donc doter les collectivités territoriales d'outils permettant de lutter contre les nuisances associées à ce trafic de transit et de favoriser la reconquête des voies structurantes des agglomérations au profit de la desserte locale et de l'intégration d'usages plus urbains, comme les transports collectifs, le covoiturage ou les modes actifs. Dans cette perspective, le présent amendement vise à autoriser l'institution d'un tarif de dissuasion du transit. Celui-ci aurait pour objet d'inciter les usagers en transit à emprunter les itinéraires dédiés de contournement des agglomérations. Un tel dispositif ne concerne que les véhicules légers, les autocars et les autobus. les poids lourds de transport de marchandises peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction de circulation sur le fondement du pouvoir de police de circulation du maire, défini par le code général des collectivités territoriales,

l'avis du Gouvernement ? Je comprends que cet amendement est initié par la métropole de Lyon pour mettre en place un mécanisme visant à écarter le trafic de transit de l'agglomération en le taxant. Le souhait d'éviter que le trafic de transit ne traverse la métropole Néanmoins, un tel dispositif, qui viserait l'ensemble des véhicules particuliers, soulève plusieurs difficultés, au-delà de la question de son acceptabilité dans le contexte actuel. D'abord, cela représente une restriction significative à la liberté de circuler.

pensons pas possible d'accompagner par des dispositions législatives, c'est la phase qui prévoirait d'observer pendant un mois

payant est un outil de régulation de la congestion et de l'occupation de l'espace dans les centres urbains. Mais il y a effectivement un principe de réalité. Dans le contexte

le trafic des camions qui se détournent d'une autoroute pour profiter des routes nationales et départementales parallèles. Je pense que c'est un vrai sujet.

dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport présentant le bilan du recueil systématique des photographies des plaques d'immatriculation des véhicules circulant sur les voies réservées. J'ai entendu que certaines demandes de rapport étaient étaient pertinentes ; je pense que c'est le cas ici. Dans son avis rendu le 15 novembre 2018, le Conseil d'État indique : « Le recueil systématique des photographies de plaques d'immatriculation des véhicules circulant sur l'ensemble des voies réservées sur le territoire national, et par conséquent, de leurs conducteurs et passagers, susceptibles ainsi d'être identifiés, est de nature à permettre la saisie sur une grande échelle de données personnelles, relatives au déplacement des individus concernés. » Le Conseil d'État ajoute par conséquent que cela peut porter atteinte au « respect du droit à la vie privée correspond également aux conclusions de la commission : « Compte tenu du caractère potentiellement intrusif pour la vie privée des conducteurs des dispositifs de contrôle, il est utile que la loi fixe des plafonds en termes de nombre de véhicules pouvant faire l'objet d'un contrôle au sein d'une ZFE. » Elle a donc adopté des amendements visant à protéger les conducteurs. La CNIL, quant à elle, n'a toujours pas rendu son avis sur la mise en place de telles dispositions. Il nous apparaît alors qu'un aperçu, même, de la situation est nécessaire. Nous regrettons la légèreté avec laquelle sont traitées les questions relatives à la collecte en masse de données alors qu'elles sont au coeur de nombreuses problématiques contemporaines. La remise d'un rapport portant sur le respect du droit à la vie privée et incluant les conclusions de cette collecte et les éventuelles mesures correctrices à y apporter nous semble donc de nature à lever les craintes légitimes exprimées de toutes parts. Quel

il est impératif de proposer aux automobilistes des solutions complémentaires permettant de réduire leur empreinte sur l'environnement. La transformation d'un véhicule à motorisation thermique en électrique, à batterie ou à pile à combustible, étant possible, une telle solution devrait être promue par les pouvoirs publics. Il s'agit en effet de répondre aux enjeux de développement durable par la mise en place d'une motorisation électrique et de s'inscrire pleinement dans une dynamique d'économie circulaire en transformant des véhicules en parfait état de marche plutôt que de les détruire. Pour rappel, en l'état du droit français, s'il est possible de transformer des véhicules vers la motorisation électrique, c'est malheureusement au prix d'une procédure complexe et coûteuse, soumise de surcroît à une demande d'accord du constructeur d'origine, ce qui est évidemment de nature à décourager toute activité industrielle et commerciale. cet amendement, nous proposons d'inscrire dans le code de l'environnement la possibilité de procéder à des transformations de véhicules à traction thermique en véhicules à traction électrique sans l'accord du constructeur, sous réserve de répondre à des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

dans des conditions définies par décret. Il s'agit de faciliter la procédure ; cela paraît effectivement souhaitable. Toutefois, je ne suis pas sûr que la suppression totale de l'accord du constructeur soit la solution pertinente. Ne conviendrait-il pas plutôt de revoir la procédure d'homologation prévue pour la simplifier ? La commission

qui pointe la lourdeur de la procédure d'autorisation par le constructeur. Pour autant, je pense qu'il faut non pas supprimer purement et simplement l'accord, mais viser à mettre en place une procédure administrative facilitée et encadrée autorisant la modification

cela a été rappelé par Patrick Chaize, la transformation d'un véhicule à motorisation thermique en véhicule électrique est techniquement possible. Peu le savent. Je l'ai moi-même appris il n'y a pas si longtemps à l'occasion d'un déplacement

au bénéfice de la planète et, bien évidemment, du pouvoir d'achat des Français. Madame la ministre, j'ai entendu la volonté qui est la vôtre de poursuivre la réflexion pour passer très rapidement à une action. Ce serait, me semble-t-il, très bénéfique pour nos concitoyens qui ont un pouvoir d'achat plus que modeste.

Il est d'une impérieuse nécessité que la lutte contre les nuisances sonores des infrastructures ferroviaires, notamment des LGV, soit menée de façon prégnante, en intégrant des indicateurs dits « événementiels » au sein de la réglementation relative aux nuisances sonores des infrastructures ferroviaires et permettant de retranscrire l'exposition de la population à des sources de bruit présentant un caractère événementiel, ce qu'on appelle les « pics de bruit En effet, dans des recommandations publiées le 10 octobre dernier, l'Organisation mondiale de la santé fait état de seuils sonores à ne pas dépasser, indiquant qu'un niveau supérieur est associé « à des effets néfastes sur la santé

et 55 décibels la nuit. Il semble donc que ces éléments ont légitimement vocation à permettre l'actualisation de l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires. Par ailleurs, nous réitérons notre volonté de voir intégrés des indicateurs « événementiels » dans le calcul des nuisances sonores en ce domaine. Pour rappel, nous avions déposé un amendement, devenu l'article 36 de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, faisant obligation au Gouvernement de rédiger un rapport d'analyse quant à l'intégration d'indicateurs dits « événementiels » dans la réglementation relative aux nuisances sonores des infrastructures ferroviaires. À la lecture de ce rapport, il est intéressant de noter, entre autres éléments, qu'une évolution de la réglementation est préconisée en fonction des pratiques et connaissances scientifiques, notamment en termes de conséquences de ces « pics de bruit » sur la santé. tenu du nombre croissant d'associations et de collectifs de riverains qui expriment leur mécontentement quant à ces nuisances sonores, nous insistons avec cet amendement sur la nécessité de réviser la réglementation en vigueur en y intégrant la notion d'émergence de bruit pour différencier les situations, élaborer élaborer des indicateurs pertinents et représentatifs du vécu des personnes et des situations réelles et en tirer les conséquences au niveau de la conception et réalisation des infrastructures. Tel est le sens de cet amendement.

la réglementation relative aux nuisances sonores des infrastructures ferroviaires n'intègre aucun indicateur de nature événementielle dans le calcul de ces nuisances, ce qui ne permet pas de retranscrire l'exposition de la population aux pics de bruit. Pour rappel, l'article 36 de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire demandait au Gouvernement la rédaction d'un rapport sur l'intégration d'indicateurs événementiels. Ce rapport préconise une évolution de la réglementation relative aux nuisances sonores des infrastructures ferroviaires selon les pratiques et les connaissances scientifiques, plus particulièrement en termes d'impact des pics de bruit sur la santé.

les situations, élaborer des indicateurs pertinents et représentatifs des situations réelles et en tirer les conséquences sur la conception et la réalisation des infrastructures.

les limites des indicateurs actuels de bruit moyen par rapport au ressenti des riverains. La nouvelle formulation est conforme aux fortes attentes exprimées par les associations de riverains, qui n'arrivent pas à obtenir une protection satisfaisante face au bruit. la Sarthe, en Mayenne et ailleurs, vous connaissez la problématique, madame la ministre : la mise en service de la LGV Paris-Rennes a profondément bouleversé la vie quotidienne des habitants de plus d'une trentaine de communes riveraines des installations ferroviaires. C'est un véritable sujet de santé publique. Ces personnes sont confrontées à des pics sonores atteignant, par moments, plus de 90 décibels, comme le reconnaît un rapport du Gouvernement remis au Parlement sur l'intégration d'indicateurs événementiels au sein de la réglementation relative aux nuisances sonores, paru en juin 2018, après l'adoption de notre amendement dans le cadre de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire.

Toutefois, la mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable n'a toujours pas rendu son rapport pourtant promis pour novembre dernier. Devant cet abandon qui laisse nos concitoyens sans solution, il est urgent de prendre des mesures qui permettent d'améliorer le cadre de vie dégradé des habitants. Cet amendement semble plus explicite que ceux de mes collègues et permettra de mieux prendre en compte les préoccupations des riverains. Quel

de trouver le bon canal pour mettre en place des procédures d'accompagnement afin de limiter les nuisances sonores. Par ailleurs, une réflexion sur les normes et la réglementation pour l'avenir